la volonté de reconnaître l'engagement de tous les soignants, y compris celui des internes et des étudiants en médecine. C'est la raison pour laquelle, dans le contexte épidémique que nous avons connu, il avait été décidé, à titre exceptionnel, que le montant des indemnités perçues au titre des gardes et des gardes supplémentaires réalisées par les externes en médecine ainsi que le montant des gardes supplémentaires effectuées par les internes seraient majorés de 50 % entre le 1 mars et le 30 avril 2020. Cela a été fait. gardes et les gardes supplémentaires effectuées par les étudiants en médecine, étant considérées comme partie intégrante de leur parcours universitaire, ne sont pas considérées comme une rémunération versée au même titre que les rémunérations salariales habituelles, ainsi que vous l'avez vous-même rappelé, monsieur le

par une difficulté rédactionnelle, puisque l'amendement renvoie sans précision au plafond mentionné au II de l'article 81 du code général des impôts. Or ce II mentionne deux plafonds distincts, ce qui peut être source de confusion. Pour ces deux raisons,

M. le rapporteur général. Monsieur le ministre, je comprends,

Je vais aller plus loin. On parle souvent de la dette qu'on laisse aux jeunes générations, de la valeur travail. J'entends que vous

Monsieur le ministre, vous allez nous faire regretter l'ancien monde, celui où Nicolas Sarkozy exonérait les heures supplémentaires ! Il ne s'agit pas là d'une rémunération. Il s'agit d'une reconnaissance envers de jeunes étudiants, qui étaient au

La possession d'une maison d'habitation en France fait partie de ces liens. Les Français non-résidents ont souvent conservé une résidence en France, où ils reviennent lors de leurs congés et où ils souhaitent s'établir en cas de retour définitif dans notre pays, notamment pour des raisons de santé, pour y prendre leur retraite ou à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou de troubles civils ou de difficultés d'emploi dans leur pays de résidence. En cette période de crise sanitaire mondiale, le souhait d'un ressortissant français de conserver une « résidence de repli » est encore plus compréhensible. Mais, depuis 2015, certaines communes peuvent appliquer une surtaxe d'habitation aux logements meublés non affectés à l'habitation principale. D'abord limité à 20 %, le taux maximal de cette surtaxe a été porté à 60 % par la loi de finances pour 2017, ce qui représente une dépense importante pour certains expatriés. C'est la raison pour laquelle, dans la proposition de loi de M. Retailleau que le Sénat a adoptée en 2019, nous avions proposé plusieurs dispositions fiscales se rapprochant de l'assimilation d'une résidence en France à une résidence principale. Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021, une trentaine de collègues députés ont déposé un amendement, dont le premier signataire était M. Frédéric Petit, visant à reprendre notre proposition sur un plan plus général. Ils ont déposé un amendement tendant à créer « une résidence de repli

nécessaire de reprendre cette proposition fondée sur l'appellation justifiée de « résidence de repli » en matière de taxe d'habitation. Nous retenons l'une des conditions prévues par l'amendement des députés : l'obligation d'être inscrit sur la liste consulaire dans le pays de résidence.

la résidence principale constitue un facteur dans l'appréciation de la domiciliation fiscale, qui ouvre ensuite droit à des avantages fiscaux. Ce que vous proposez pourrait donc s'avérer extrêmement coûteux.

que les projets de loi de finances rectificative devaient comporter le moins de dispositions fiscales possible, convaincus que la stabilité fiscale nécessitait plutôt des dispositions votées en fin d'année pour une application à +1 et que les PLFR avaient avant tout comme objectif de redéployer ou de déployer des crédits en fonction des besoins de fin de gestion ou des réponses à la crise. Dans ce PLFR, quelques dispositions fiscales s'inscrivent uniquement

de supprimer la surtaxe pour les résidences de repli des résidents à l'étranger. Quel

est à M. Éric Bocquet. Monsieur le ministre, vous nous aviez confié, lors de l'examen du PLF pour 2021, que nous avions oublié des types de revenus générés par les sociétés d'investissement immobilier cotées. Vous avez cette qualité appréciable d'écouter les parlementaires. Pour notre part, nous vous avons si bien écouté que nous vous proposons ici de revenir sur l'exonération d'impôt sur les sociétés dû par les SIIC pour les exercices 2020 et 2021.

pour ensuite prendre des mesures de soutien aux petits commerces et aux entreprises en difficulté. Voilà le sens de la redistribution et le sens de l'impôt ! Les grandes foncières se portent bien. Pour vous donner quelques chiffres, elles ont servi un rendement d'environ 6 % brut sur sur la base de leurs dividendes en cours en 2019, soit environ 4 % net après imposition à la de 30 %. est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à augmenter le taux de l'impôt sur le revenu pour les années 2020 et 2021 pour les revenus tirés des

défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Si nous nous sommes écoutés, monsieur Bocquet, nous ne nous sommes pas nécessairement tout à fait compris sur les objectifs. D'abord, nous avons privilégié d'autres mesures pour accompagner les entreprises que vous souhaitez aider par ce type de dispositif. Je pense notamment à la défiscalisation des abandons de créances de loyer, qui a par ailleurs été prolongée à l'occasion de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. J'ajoute que les sociétés mentionnées 1655 du code général des impôts, auquel vous faites référence, correspondent aux sociétés immobilières de copropriété et non pas aux SIIC que vous visez dans l'objet de l'amendement. Ensuite, l'article 187 du CGI s'applique aux seuls actionnaires non-résidents, de sorte que votre amendement ne permettrait pas de toucher l'ensemble des actionnaires des SIIC, contrairement à ce que vous souhaitez. Ces deux difficultés de forme s'ajoutent à la préférence que nous avons eue pour d'autres modalités d'accompagnement des entreprises.

Le régime fiscal des donations est aujourd'hui soumis à une contrainte d'âge pesant sur le donateur, qui doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation. Cette contrainte freine largement la circulation du capital entre les générations. Compte tenu de l'allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles, qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par le rehaussement de l'âge maximal du donateur de 80 à 90 ans. Cette mesure paraît d'autant plus pertinente qu'une forte épargne a été accumulée pendant la crise et que les jeunes générations pourraient être plus promptes à dépenser et à investir cette épargne à la faveur de la relance de l'économie.

savez, la limite d'âge à 80 ans est une mesure anti-abus pour faire en sorte que les dons de sommes d'argent consentis en franchise d'impôt ne donnent pas lieu à une optimisation fiscale par trop débridée. Je rappelle que l'âge de 80 ans est globalement proche aujourd'hui de l'espérance de vie moyenne.

afin que le patrimoine soit plus facilement transmis aux jeunes actifs au moment où ceux-ci en ont le plus besoin. Il tend à porter l'abattement applicable aux donations à 100 000 euros. La

avons déjà adopté, sur l'initiative du Sénat, un dispositif permettant, pour une durée temporaire- du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 -, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les dons versés en numéraire jusqu'à 100 000 euros. Par ailleurs, le dispositif prévu par ces amendements ne prévoit aucune condition de réemploi dans des activités favorables à l'économie.

Les exonérations et abattements de droit commun sont actuellement très favorables. Par exemple, en cumulant l'abattement spécifique aux petits-enfants d'un peu plus de 30 000 euros et l'exonération des dons familiaux de même montant, deux grands-parents de soixante-quinze ans peuvent d'ores et déjà donner à chacun de leurs quatre petits-enfants jusqu'à presque 127 500 euros

Or, on le sait, avec les prix de l'immobilier, créer une famille à Paris ou dans une métropole est très difficile. Les jeunes ont besoin de cash pour pouvoir s'installer. Je voterai donc ces amendements.

au 31 décembre 2022,

des impôts, la donation entre parents, sans droits et sans conditions d'usage, d'un montant de 50 000 euros maximum.

C'est pourquoi nous revenons également avec cet amendement visant à instaurer un impôt sur la fortune fondé sur l'empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 800 000 euros. Le Haut Conseil pour le climat rappelait hier que les deux tiers des Français- et pas les plus riches ! - sont fortement ou très fortement impactés par le dérèglement climatique. Nous ne subissons pas tous de la même manière les inégalités climatiques

le plus. En France, l'empreinte carbone moyenne d'un individu appartenant aux 10 % les plus riches est de 17,8 tonnes de CO2 par an, contre seulement 3,9 tonnes pour les 50 % les plus pauvres.

! Monsieur le ministre, ce matin, le Conseil d'État vous a donné neuf mois pour adopter des mesures supplémentaires permettant de respecter l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Je vous le demande, ne serait-ce pas le moment, grâce à ces propositions, notamment

a d'ailleurs remis un rapport le 1 octobre 2019 dans lequel il est indiqué que les gains fiscaux issus de la mise en place de la se sont concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés, plus particulièrement sur les 5 % les plus aisés. Ces derniers ont ainsi bénéficié en 2018 d'un cadeau fiscal de 1 000 euros en moyenne. Une fois encore, la stratégie budgétaire et fiscale du Gouvernement est bien celle d'un soutien aux très riches, alors même que la théorie fumeuse du ruissellement est jour après jour toujours plus discréditée. La seule hypothèse crédible d'un point de vue économique et politique demeure une taxation juste du capital, ce qui n'est clairement plus le cas depuis 2017. Tel est l'objet du présent amendement.

sont captés par 1,7 % des foyers fiscaux. La concentration est encore plus forte quand on progresse dans la hiérarchie des déciles : 0,1 % des foyers accaparent les deux tiers des dividendes, un tiers étant même empoché par 37 000 foyers, sur 38 millions de foyers fiscaux que compte notre pays. L'Institut des politiques publiques est d'avis que le dispositif est « peu susceptible de conduire à une hausse de l'investissement privé ». Tel est le sens de cet amendement.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à mettre fin à la familiarisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et à augmenter ses taux. Créée par Nicolas Sarkozy au lendemain de la crise de 2008, cette contribution est un élément de la participation des hauts revenus au financement de la crise. Nous proposons de l'élargir.

de la population.

Aussi, 40 % des Français épargnent en moyenne moins de 5 %, quand les 20 % des plus aisés épargnent 28 % de leurs revenus. En valeur, les 20 % épargnent quinze fois plus que 40 % des Françaises et des Français.

: réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme, et réduire ainsi les risques d'instabilité. Les politiques menées s'accompagnent d'une augmentation permanente de la valeur des actifs,

Ces moyens pourraient venir financer des politiques publiques en matière de solidarité internationale, notamment en matière d'aide publique au développement Compte tenu du contexte sanitaire actuel, singulièrement pour l'Afrique, l'engagement présidentiel de porter l'APD à 0,55 % du PIB en fin de mandature doit trouver une traduction concrète dès cette année, afin de lutter efficacement contre la pandémie. Au surplus, nul ne peut contester les besoins de financement des vaccins dans les pays en voie de développement, qui nécessitent une réponse ferme de la France. Aussi, dans un souci de responsabilité, les auteurs de cet amendement veulent simplement aider le Gouvernement à tenir ses promesses.

Mme Isabelle Briquet. Le présent amendement vise à moduler le mécanisme de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages, qui est organisé par l'article 235 X du code général des impôts. La baisse de l'accidentologie et de la sinistralité du fait de la crise sanitaire est telle qu'il paraît tout à fait opportun d'appeler les acteurs de l'assurance à assumer leurs responsabilités et à contribuer à l'effort national pour redresser le pays. Après deux confinements, les assurances ont réalisé de substantielles économies, notamment sur leurs contrats automobiles. Si les chiffres divergent selon les interlocuteurs, ils sont tout de même éloquents. Lors du premier confinement et pour la seule assurance automobile, le cabinet Addactis a estimé, à la fin du mois d'avril 2020, que les compagnies d'assurances économiseraient près de 1,5 milliard Ces estimations ont même été revues à la hausse dans une nouvelle étude du 7 mai : la baisse de la sinistralité automobile pourrait atteindre jusqu'à 80 % pendant la période de confinement. Plus de 2,2 milliards d'euros sont évoqués, selon l'association UFC-Que Choisir. mi-septembre, un rapport du Gouvernement remis au Parlement est venu étayer ces données, en évaluant, sur la base des retours volontaires des compagnies d'assurances, à moins 38 % l'évolution des sinistres automobiles payés entre avril-mai 2019 et avril-mai 2020

de compter sur les acteurs qui ont aujourd'hui la capacité de le faire. Le mécanisme proposé vise à taxer les excédents des provisions au moment où ils sont réintégrés dans leurs résultats par les entreprises d'assurances. Il est parfaitement possible à ces acteurs de sortir de leurs résultats les moyens financiers mis de côté en vue du paiement de l'indemnisation. Il est alors appliqué un taux d'intérêt à cette réintégration, afin d'éviter un effet d'aubaine et de traiter les sommes provisionnées de façon excessive, comme si elles avaient dû être acquittées au moment de leur provisionnement. Il est donc proposé de faire passer le taux mensuel d'intérêt de 0,40 % à 0,50 % en 2021, puis à 0,60 % à compter de Le contexte actuel, extraordinaire, peut conduire les entreprises d'assurances à surprovisionner, à la suite d'une sinistralité 2020 particulièrement sujette à plonger, faute de garanties dues contractuellement, avec l'immobilisation des Français en raison du confinement.

la pandémie, à un moment où, ici même, nous avions fait pression sur le monde de l'assurance. Pour être tout à fait objectif, je rappelle que le secteur de l'assurance est le seul au financement de la crise à hauteur de 400 millions d'euros, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué de créer un certain nombre de tensions. En effet, il ne vous aura pas échappé que les acteurs, selon leur forme capitalistique ou mutualiste,

composé en quasi-totalité de TPE et de PME, de survivre. Ses acteurs se sont mobilisés afin d'adapter leur représentation à un cadre sanitaire viable.

de tenir compte de cette situation particulière. Le nombre de représentations nécessaire pour être éligible au dispositif a ainsi été ramené de quatre à deux, le nombre de lieux de représentation de trois

au dispositif d'activité partielle et au PGE, dont a aussi bénéficié le secteur. Dans le cadre de ce PLFR, nous inscrivons 150 millions d'euros de crédits complémentaires, dont une part importante consacrée au spectacle vivant,

: La parole est à Mme Monique de Marco. Le secteur des transports est responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Il doit davantage évoluer et s'adapter aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux, notamment en accompagnant des activités comme le rétrofit,

L'étude de l'Ademe de mai 2021 démontre que le rétrofit électrique est une solution convaincante pour les enjeux de qualité de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre. Le rétrofit électrique permet le réemploi de la carcasse du véhicule thermique déjà en circulation. Par rapport à un véhicule neuf, il évite la fabrication de nouvelles carcasses et les émissions de gaz à effet de serre associées. Enfin, en tant que véhicule électrique, le véhicule rétrofité évite les rejets de polluants atmosphériques et d'échappement lors de sa phase d'usage. Par ailleurs, la filière du rétrofit électrique est pourvoyeuse d'une activité pouvant consolider des emplois non délocalisables. L'électrification progressive du parc de véhicules ira naturellement de pair avec une baisse des activités d'entretien et de maintenance des garagistes, puisque le véhicule électrique nécessite moins d'entretien qu'un véhicule thermique. En ce sens, le rétrofit pourrait permettre à la filière de se renouveler et de conserver un maximum d'emplois locaux.

Pour les plus rurales d'entre elles, à faible potentiel fiscal, c'est une charge financière importante qui est devenue « incompressible ». Le présent amendement vise à rétablir l'éligibilité de ces dépenses au FCTVA. La

des dépenses exposées par les communes et leurs EPCI pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme, ainsi que pour la numérisation du cadastre. La modification introduite dans la loi de finances pour 2021, à l'article 251, 251, a un impact direct et financier sur les communes, sur les communautés de communes ayant pour compétence l'élaboration des PLUi, ainsi que sur les établissements publics porteurs de SCoT. Plus largement, l'ensemble des collectivités chargées de la compétence « urbanisme » à l'échelle nationale sont concernées. Aussi, le présent amendement vise à modifier l'article L. 132-16 du code de l'urbanisme pour revenir à la situation antérieure.

pour toutes dépenses imputées sur un des comptes visés par un arrêté ministériel. Cette réforme entraîne des modifications de l'assiette des dépenses éligibles et, par suite, suscite des inquiétudes bien légitimes, notamment celles que vous avez évoquées concernant les documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre.

La suppression de ces montants perçus par les EPCI à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021. Cependant, la compensation de référence de taxe d'habitation sur les résidences principales prendra en compte, entre autres éléments, le taux de taxe En fin de dernier mandat, certaines équipes intercommunales s'étaient engagées à mettre en place des pactes financiers et fiscaux territoriaux. En effet, la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine avait conféré un caractère obligatoire à ces pactes financiers dans les communautés signataires d'un contrat de ville. L'année 2017 a finalement été retenue comme année de référence pour la compensation. Ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement alors même qu'elles ont fait preuve de volontarisme et de sérieux prospectif dans leur organisation financière Afin de ne pas pénaliser les EPCI qui ont adopté des pactes financiers et fiscaux avant 2019, le présent amendement tend à fixer à 2018, au lieu de 2017, l'année de référence dans le calcul du montant de la taxe d'habitation. Quel de la commission ? Vous proposez que, dans le cas où un EPCI et ses communes membres ont conclu un pacte financier et fiscal se traduisant par une modulation des taux communautaire et communal de la le taux intercommunal de référence pour le calcul des compensations soit celui de l'année 2018. Je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons. Tout d'abord, sur le plan technique, plan technique, il ne va pas au bout de sa logique et omet de prévoir, notamment, une minoration à due concurrence des compensations perçues par les communes. En effet, dans la situation que cherche à résoudre cet amendement, si le taux intercommunal a augmenté entre 2017 et 2018, c'est que le taux communal a diminué d'autant. En conséquence, les compensations au profit des communes devraient être calculées sur la base d'un taux plus faible. Ensuite, sur le plan pratique, les EPCI et leurs communes membres disposent, à mon sens, de tous les leviers budgétaires permettant de rétablir l'équilibre financier auquel ils étaient parvenus. Cela peut passer, par exemple, par une modulation des dotations de solidarités communautaires ou par l'ouverture de fonds de concours. À compter de 2023, on peut même envisager que les taux des impôts fonciers soient rééquilibrés entre l'EPCI et ses communes.

qui ont fait le choix de baisser les impôts entre 2017 et 2018 : l'application des dispositions proposées conduirait automatiquement à une baisse de la compensation qu'elles perçoivent.

Si la contribution à l'audiovisuel public s'établit à environ 3,2 milliards d'euros, dont 118 millions d'euros proviennent des comptes professionnels, tous secteurs d'activité confondus, cette exonération représenterait au final 20 millions d'euros. Ce serait une économie bienvenue pour l'ensemble de ces établissements, qui ont énormément souffert de la crise liée tient à ce que cette nouvelle mesure de soutien occulte celles déjà mises en oeuvre en faveur de la trésorerie des entreprises de ce secteur. La seconde tient à l'absence d'égalité de situation entre les entreprises concernées : l'hôtellerie n'a pas été directement impactée par les mesures de fermeture ; les cafés et les restaurants, eux, ont pu rouvrir avant la fin du premier semestre, à la différence des établissements de nuit. Dans ces conditions, une réduction de moitié de la contribution à l'audiovisuel public ne paraît pas conforme à la réalité de l'usage des téléviseurs selon le type d'établissement. C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

de TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour le gazole non routier, le

Au total, les dépenses fiscales relatives au carburant représenteraient 2,4 milliards d'euros de perte de recettes pour l'État ; or c'est aussi une aide apportée aux entreprises industrielles et agricoles, au secteur du bâtiment et travaux publics, ainsi qu'au transport ferroviaire non électrifié. M. le rapporteur général

janvier 2023 et non au 1 juillet 2022 l'alignement du tarif de TICPE applicable au GNR sur celui du gazole routier. Il est nécessaire de tenir compte du contexte économique dégradé en raison de la crise sanitaire. Le secteur du bâtiment et des travaux publics a été fragilisé par les conséquences de cette crise sanitaire : situation de leur

devait s'aligner progressivement sur la fiscalité du gazole routier, sauf pour les engins agricoles. Les professionnels bénéficient jusqu'ici d'un avantage fiscal qui consiste en un tarif réduit de TICPE.

2022. Les députés ont adopté un amendement visant à reporter d'un an cette hausse et à supprimer la niche fiscale en une seule fois, le 1 juillet 2021. Mais, par le biais d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité reporter encore une fois cette hausse de dix-huit mois, jusqu'à janvier 2023.

La crise sanitaire ne doit pas exempter les entreprises, en particulier dans les secteurs du transport et du BTP, de faire les efforts nécessaires pour adapter leurs activités au réchauffement climatique. Le rôle de l'État et notre rôle sont bien d'accompagner les acteurs, mais pas de renoncer à agir.

Cette niche fiscale est coûteuse pour les finances publiques et son efficacité économique paraît relativement faible. Elle est également coûteuse, cela a été rappelé, pour l'environnement. Il s'agirait, bien sûr, de mettre en place un dispositif d'accompagnement nécessaire des entreprises concernées, mais par d'autres moyens. Il faut y réfléchir. Nous proposons donc la suppression de cet article 2 pour mettre fin au cycle incessant des reports.

Par ailleurs et de façon plus discrète, au détour d'un article dont l'ensemble des implications sont difficiles à analyser par des non-initiés, le Gouvernement a prévu de supprimer des mesures d'équité et de lutte contre la fraude qui avaient été adoptées par le Parlement à l'occasion du projet Ces mesures ont vocation à prévenir les risques de concurrence déloyale liés à la réalisation des travaux relevant du BTP par des personnes qui exercent à titre principal une activité agricole et qui continueront, à ce titre, à avoir accès à un carburant à tarif réduit. Elles prévoient notamment la création d'un carburant coloré spécifique à l'activité du bâtiment, ainsi que l'établissement d'une liste d'engins susceptibles de recourir aux carburants agricoles.

celle du maintien dans la loi des dispositifs d'accompagnement sur lesquels le Gouvernement s'était engagé. L'amendement que je porterai au nom de la commission visera, d'une part, à rétablir la date du report au 1 janvier 2023 d'autre part, à maintenir dans la loi les deux dispositifs d'accompagnement auxquels les acteurs économiques sont le plus attachés : le gazole BTP et l'arrêté dressant la liste d'engins.

à rétablir le gazole BTP et la liste d'engins. Je précise qu'un alinéa de l'article 265 du code des douanes, lui aussi supprimé, prévoyait la création d'un registre obligatoire de travaux, susceptible de faciliter les contrôles de l'administration sur l'utilisation du gazole agricole. Ce dispositif, qui n'est pas véritablement souhaité par les professionnels du BTP, entraînerait

que la date d'entrée en vigueur d'une réforme est repoussée, il n'y a pas lieu de mettre en place les mesures de contrôle en avance de phase. J'indique, par ailleurs, indépendamment de l'avis que je donne à cet instant, que nous avons créé un dispositif de suramortissement pour les travaux publics dans le cadre de la mise en oeuvre de cette réforme, lequel dispositif n'est pas supprimé ; et nous n'en proposons pas la suppression.

Effectivement, le sujet du gazole non routier revient dans les hémicycles du Parlement français ... Ce sujet préoccupe de longue date nos entrepreneurs de travaux publics et du paysage, que nous recevons très fréquemment dans nos permanences. Ils font des efforts et aimeraient bien décarboner leurs outils de travail, mais il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Il faut donc bien les accompagner ! Le débat qui nous occupe concerne aussi le respect de la parole publique. Les représentants de ces entreprises étaient sur le point de faire une grande manifestation

comme l'avait dit votre prédécesseur Gérald Darmanin lors de l'introduction de cette nouvelle tarification à l'Assemblée nationale le 17 décembre 2019. Cet alinéa ouvrait donc la possibilité de produire un carburant avec une nouvelle couleur « spéciale BTP non routier afin de sécuriser l'application du remboursement agricole de la TICPE, selon les termes de l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental. Si des difficultés techniques et opérationnelles ont pu être soulevées, c'est que le délai initial d'application de la loi était fixé au 1 juillet 2020, ce qui laissait effectivement peu de temps, c'est-à-dire six mois, pour sa mise en oeuvre, avec un report de deux ou trois mois en fonction de l'avancée de nos discussions. Cet argument ne tient plus.

Compte tenu du contexte économique et des difficultés que rencontrent actuellement les acteurs du bâtiment et des travaux publics du fait des tensions constatées dans l'approvisionnement des matières premières, le Gouvernement a décidé de reporter au 1 janvier 2023 l'entrée en vigueur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

est à M. Éric Bocquet. Alors que, pendant près de deux semaines, le Sénat, à la suite de l'Assemblée nationale, s'est penché sur le projet de loi Climat, il ne s'est pas donné les moyens de son ambition rehaussée, comme l'explique le média.

les mesures qu'il contient ne permettront pas d'atteindre cet objectif ambitieux. On peut toujours chercher les bonnes raisons de retarder l'échéance, mais vous ne trouverez que de mauvaises raisons pour vous dédouaner de vos responsabilités au regard de la catastrophe climatique de plus en plus présente et pressante.

Dans ce cadre, la suppression de la politique fiscale accommodante- ou, pour le dire autrement, la suppression de la niche fiscale dont bénéficie le transport aérien, notamment le fret aérien, fortement émetteur de gaz à effet de serre -serait logique.

Chaque fois que nous déposons cet amendement, on nous rétorque systématiquement que la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale de 1944 exempte de toute taxe les carburants d'aviation destinés aux vols internationaux. Cependant, la directive 2003/96/CE du Conseil prévoit que les États membres peuvent limiter son champ d'application aux transports internationaux et intracommunautaires, ce qui signifie que la taxation des seuls vols nationaux est donc bien possible et que rien ne s'oppose à ce que l'on rétablisse pour eux

infra ou intra-européens ne sont pas tous en faveur de la France. Il faut donc être vigilants et ne pas se mettre trop vite des boulets aux pieds.

La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet le transport ferroviaire, avec pour conséquence un effondrement des recettes pour la SNCF ; s'y ajoutent les conséquences du mouvement social contre la réforme des retraites. S'il n'est pas question de remettre en cause l'effort budgétaire significatif opéré lors du plan de relance, à hauteur de 4,7 milliards d'euros, le groupe socialiste a très tôt dit qu'il ne serait pas suffisant pour remettre l'entreprise à flot et, dans le même temps, lui permettre d'investir massivement. Cet amendement s'inscrit donc dans l'ensemble des propositions faites par le groupe socialiste depuis plusieurs années, et encore récemment dans le cadre de la loi Climat et résilience, visant à affirmer le principe « pollueur-payeur » : les secteurs les moins vertueux doivent être davantage mis à contribution que les autres. Parce qu'il s'agit d'un secteur clé pour la réussite de la transition écologique, qu'il faut fortement accompagner, soutenir et développer à court, moyen et long terme, les auteurs de l'amendement proposent, en sus des efforts budgétaires précédemment cités, de supprimer la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires et la contribution de solidarité territoriale, des impôts de production dont les seules entreprises ferroviaires sont redevables.

La suppression de ces contributions ne doit pas entraîner pour autant la suppression du soutien au développement des trains d'équilibre du territoire, tel qu'initialement prévu par le compte d'affectation spéciale. Au contraire, il s'agit de contribuer à la compétitivité de l'ensemble du secteur ferroviaire vis-à-vis de ses concurrents moins vertueux écologiquement, tant pour la mobilité des personnes que pour celle des marchandises. Le groupe socialiste salue le rapport de trains d'équilibre du territoire, présenté il y a quelques semaines, et attend avec impatience la présentation de la stratégie fret du Gouvernement, qui doit avoir lieu dans les prochaines semaines.

des résultats de l'opérateur assujetti, c'est-à-dire la SNCF. Or, du fait de la perte d'activité très forte de l'année 2020, en 2021, la contribution que vous proposez de supprimer sera extrêmement basse par rapport aux 242 millions d'euros affichés dans le projet de loi de finances pour 2020. Nous estimons qu'elle passerait de 242 millions à moins de 20 millions d'euros.

ces deux éléments de fiscalité, qui contribuent au développement des trains d'équilibre du territoire. Notre objectif, dans le cadre de l'ouverture progressive à la concurrence du fret comme du transport de voyageurs, est d'abaisser le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel les opérateurs concurrents de l'opérateur historique seront assujettis à ces deux contributions. Cela permettra de rétablir l'égalité entre l'opérateur historique et ses éventuels concurrents, sans enlever à l'État

La taxe sur l'aviation civile est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) considère qu'une unité de trafic correspond à un passager ou à 100 kilos de fret, soit 0,1 tonne. Pourtant, le niveau de la taxe sur l'aviation civile ne respecte pas ce principe. En effet, un passager, soit une unité de trafic, paie entre 4,63 euros de taxe pour un vol intra Union européenne et 8,32 euros pour toute autre destination, tandis qu'une tonne de fret, soit dix unités de trafic, est actuellement taxée à 1,38 euro. Cette absence de proportion équivaut à une niche fiscale hautement contestable accordée au fret aérien, sans justification. Le fonctionnement du transport aérien doit être amélioré, car ce secteur contribue beaucoup, eu beaucoup, eu égard à son tonnage, à la pollution atmosphérique et à l'augmentation des gaz à effet de serre, en raison en particulier des exonérations dont il bénéficie. Il faut agir ! Alors, j'entends bien, monsieur le rapporteur général, que tout va toujours trop vite et qu'il faut toujours attendre,

du désarroi, parce que votre logique politique libérale n'est en réalité, on le voit, pas compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique.

D'abord, je rappelle que le produit des amendes de police, vous le savez, n'est ni un produit fiscal ni un produit domanial, ce qui l'exclut à nos yeux du filet de sécurité. Ensuite, la répartition de ce produit s'opère en faisant une distinction en fonction de la taille des collectivités, alors que toutes les collectivités locales bénéficient pareillement du filet de sécurité. Enfin, la recette est affectée à la section d'investissement et non à la section de fonctionnement, ce qui ajoute un élément de complexité. Cela étant, la situation conjoncturelle très particulière

de rebudgétisation. Celle-ci permettrait de garantir un produit qui soit le plus stable possible, indépendamment du niveau de recettes obtenues par l'État la mise en place des amendes et des timbres-amendes. Cela fait partie des pistes sur lesquelles nous travaillons, et je forme moi aussi le voeu que nous puissions aboutir d'ici au prochain PLF de manière à avoir plus de lisibilité et de prévisibilité sur ce poste de recettes pour les collectivités locales.

2020, n'ayant pas pu présenter d'amendements, comme le rappelait Christine Lavarde, du fait des règles de la LOLF. Nous n'avions pas non plus obtenu de réponse du ministre.

pour Île-de-France Mobilités. À la suite d'un nouvel amendement du rapporteur général à l'Assemblée nationale, ce PLFR prolonge le dispositif d'avance remboursable pour faire face à l'effondrement des recettes d'Île-de-France Mobilités pendant les

entre le mécanisme de filet de sécurité sur les pertes de recettes tarifaires et celui de l'avance remboursable d'un peu plus de 1 milliard d'euros au titre des pertes de recettes tarifaires. Je demande le retrait de l'amendement.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a voté l'intégration d'IDFM dans le filet de sécurité pour les recettes fiscales au cours de l'année 2021, ce qui est une protection supplémentaire. L'avis est défavorable.

régionales ... Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, disait qu'il fallait trouver un meilleur équilibre et des compensations réelles par rapport aux pertes très lourdes d'IDFM en 2020-2021. Je comprends très bien que vous n'ayez pas de réserve d'or à Bercy et que vous ne puissiez pas faire beaucoup d'avance, mais de là à dire qu'on a trouvé une solution

je doute que la RATP et la SNCF Île-de-France puissent continuer de fonctionner de manière normale, avec des investissements normaux et des matériels nouveaux, si l'État ne fait pas un effort de compensation. La vote. Je remercie Roger Karoutchi de son intervention, qui me paraît relever d'un certain bon sens. L'année dernière, la majorité sénatoriale avait accepté l'avance remboursable, depuis, il y a eu de nouvelles périodes de confinement. Disposer d'un filet de sécurité sur les recettes fiscales mais pas d'une véritable compensation et d'une vraie prise en charge des pertes de recettes tarifaires, cela ne me paraît pas raisonnable.

ou d'en diminuer le taux. Cette mesure est pleine de bon sens, car elle encourage la mise en place d'une agriculture respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Néanmoins, elle est particulièrement difficile à mettre en place dans les communes ayant peu de ressources, comme les plus petites d'entre elles. En effet, leur budget restreint est souvent trop difficile à équilibrer pour permettre de mettre en place l'exonération de la taxe foncière pour les agriculteurs qui se convertissent au bio. Dès lors, cet amendement vise à ce que le manque à gagner pour ces petites communes qui mettent en place cette exonération de taxe foncière soit intégralement compensé par l'État. Ce serait une manière de répartir l'effort et cela bénéficierait, à terme, à la préservation Pour information, cet amendement a le même objet que l'amendement suivant de Mme Delattre.

Je précise par ailleurs que l'amendement ne me paraît pas opérant, puisqu'il vise à ce que cette compensation se traduise par une majoration globale de la DGF, qui est répartie entre les collectivités selon des modalités propres. La DGF supplémentaire qui reviendrait aux communes et EPCI ne correspondrait donc pas au coût de l'exonération décidée. L'avis est défavorable.

la cible ne sera probablement pas atteinte. Il convient donc d'encourager un peu plus le soutien à l'agriculture biologique. Au-delà des soutiens mis en oeuvre au travers de la PAC, l'agriculteur peut solliciter une exonération du paiement ou une diminution du taux de sa taxe foncière en contrepartie de la conversion de son exploitation au bio. Si ce levier apparaît opportun sur le principe, il entraîne bien entendu un manque à gagner budgétaire pour les communes du fait de la non-compensation dispositif. Aussi, les petites communes, qui ont des budgets serrés, se voient, hélas ! contraintes de refuser cette aide à leurs agriculteurs, afin de ne pas fragiliser leurs finances et pénaliser d'autres politiques locales. L'amendement vise donc à augmenter de 1 million d'euros le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Plus directement, monsieur le ministre, comment soutenir les communes qui souhaitent encourager les pratiques vertueuses en agriculture ?

des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte. Le PLFR pour 2020 prévoit que la dotation s'applique aux pertes de recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation. Cet amendement ajoute à cette liste la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation, dont les produits sont également affectés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

d'outre-mer et à la collectivité de Corse. Cette garantie, qui se traduit par une dotation versée sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, porte sur des recettes fortement sensibles à la conjoncture. Le dispositif proposé permet donc d'assurer un traitement égal de l'ensemble des collectivités concernées par ces dispositifs et de donner aux élus locaux la meilleure visibilité possible sur l'évolution de leurs ressources.